et vous nous avez dit, l'an dernier, que le budget pour 2019 s'inscrivait dans la continuité du précédent. Au sein de ces deux budgets, nous n'avions pu trouver aucune nouveauté répondant aux grands enjeux que doit relever l'agriculture française, et nous nous étions abstenus, considérant que l'essentiel restait à faire. Dans notre démocratie, l'acte politique majeur est le vote du budget, et c'est à l'aune des difficultés et des grands enjeux de transformation auxquels l'agriculture de notre pays est confrontée que le budget présenté aujourd'hui par le Gouvernement doit être apprécié. Le revenu des agriculteurs, l'accompagnement de la transformation agroécologique des exploitations, la compétitivité des filières, la gestion des risques, le budget et la gouvernance de la future PAC, la stratégie politique en faveur de la forêt et de la filière bois, l'anticipation des conséquences du Brexit pour la pêche : voilà les sujets sur lesquels notre appréciation doit porter. Pour ce qui est du revenu agricole, l'évaluation des premiers effets de la loi Égalim par nos collègues rapporteurs fait apparaître, à mi-parcours de l'expérimentation et du point de vue des producteurs, une inefficacité totale.

Il y a trois ans, avec Henri Cabanel et vous-même, monsieur le ministre, nous avions ensemble fait voter à l'unanimité du Sénat un texte relatif au développement des outils de gestion des risques en agriculture. Nous proposions même la mise en place, dans le cadre des règlements européens, d'un fonds de stabilisation du revenu agricole. Ce texte n'a pas alors été repris par l'Assemblée nationale, mais il pourrait certainement l'être aujourd'hui, sur votre initiative. le règlement européen Omnibus a été adopté ; il assouplit les mécanismes de gestion de ces fonds de mutualisation des risques et d'éligibilité à ceux-ci. L'État est bien entendu partie prenante à ces financements, mais rien dans le budget ne semble avoir été prévu pour déployer ces dispositifs,

je peux vous dire, pour avoir rencontré leurs représentants il y a quelques jours, que les filières sont extrêmement inquiètes des déséquilibres qui apparaissent sur certains marchés et des conséquences de la surtaxation par les États-Unis de nos produits d'exportation.

n'avaient pas besoin de cela ! Vous envoyez là un signe contredisant l'intention initiale de redonner du revenu aux producteurs. Maintenir ce dispositif est indispensable, quand bien même des allégements de charges s'y ajoutent. Je regrette que l'amendement de préservation intégrale du dispositif que nous avions présenté lors de l'examen du PLFSS n'ait pas été adopté. La compétitivité des filières concernées ne s'en serait que mieux portée, dans ce contexte de guerre économico-diplomatique, auquel s'ajoute en permanence une compétition sur les coûts de production. La transition agroécologique vers des produits de qualité à prix abordables en serait aussi facilitée. Nous savons tous ici que la fin de l'utilisation du glyphosate et la création de zones de non-traitement vont se traduire par des surcoûts de production de l'ordre de 50 à 150 euros, voire plus,

Par conséquent, nous proposerons un amendement de création d'un « fonds spécifique d'aide et d'accompagnement à l'arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires », doté de 10 millions d'euros.

C'est le cas dans le Gers, pour près de 110 éleveurs, dans l'Aude, dans les Deux-Sèvres, ailleurs aussi. Nous ne pouvons toujours pas l'admettre, nous qui connaissons les territoires concernés, les hommes et les femmes qui y vivent avec autant de peine que de dignité Pour faire face à ces baisses de revenus, nous pensons qu'il serait judicieux de développer expérimentalement des paiements pour services environnementaux (PSE) sur ces territoires.

du premier pilier, du second, dont les territoires ruraux vont aussi probablement faire les frais, ou du « verdissement », dont l'accompagnement pourrait être sensiblement amoindri, ce qui retardera d'autant la transition vers un modèle durable d'agriculture. d'ores et déjà que le Brexit aura une incidence sensible sur le budget de la PAC. La pêche est, à cet égard, un autre sujet particulièrement préoccupant, qui nécessite d'anticiper. La politique déployée en matière de forêts et de soutien à la filière bois ne nous paraît pas non plus adaptée aux enjeux et au potentiel de notre pays.

Il faut en outre donner à l'agriculture dite endogène d'outre-mer les moyens de son développement ; nous proposerons d'y affecter 5 millions d'euros. Monsieur le ministre, malgré une hausse faciale de 400 millions d'euros à périmètre constant, ce budget pour 2020 ne prend pas ou pas assez en compte les grandes difficultés des filières,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je concentrerai mon propos sur la filière forêt-bois, plus vulnérable que jamais. Plusieurs effets se conjuguent pour fragiliser nos forêts, qui meurent, si j'ose dire, « à petit feu sécheresses à répétition, fortes chaleurs, attaques parasitaires, dégâts de gibiers croissants ... Plus aucun territoire, plus aucune essence ne sont épargnés. À la catastrophe écologique s'ajoute la menace économique : des communes forestières privées de ressources, des marchés saturés,

à devenir plus résilientes, en privilégiant des essences plus résistantes à la chaleur et plus frugales en eau, en diversifiant les peuplements, en faisant évoluer les méthodes sylvicoles, mais aussi en innovant et en adaptant l'outil de transformation. De nombreux pays ont compris l'intérêt d'une forêt régénérée, productrice de bois d'oeuvre et d'énergie renouvelable et puits de carbone : certains de nos voisins européens, mais aussi la Chine, la Russie ou l'Australie, investissent massivement dans leurs forêts. La France, pourtant riche d'une forêt multifonctionnelle de 17 millions d'hectares, source de plus de 400 000 emplois, ne considère pas encore sa ressource forestière à la hauteur de ses bienfaits. Cette négligence se traduit dans le PLF pour 2020 : le Gouvernement prévoit une baisse de 2,5 % des crédits. crédits destinés à la forêt publique, l'Office national des forêts (ONF), sont maintenus, il n'en est pas de même pour la forêt privée, qui représente pourtant les deux tiers des surfaces forestières. Le Centre national de la propriété forestière perd 1 million d'euros, soit 7 % de son budget. Comment, dès lors, assurer sa présence et la disponibilité des 451 équivalents temps plein actuellement en service, qui ne sont pas de trop sur le terrain, aux côtés des 3 millions de propriétaires ?

18,5 millions d'euros est affectée au fonds stratégique de la forêt et du bois. C'est moins qu'à sa création, en 2014. Il était alors doté de 25 millions d'euros, et devait atteindre les 100 millions Aujourd'hui, les sylviculteurs craignent de devenir à leur tour les victimes d'un « sylvi-bashing » condamnant sans discernement les méthodes d'une profession pourtant exemplaire, qui pratique la multifonctionnalité, le mélange des essences, le respect des cycles et des sols, plus que dans tout autre pays au monde C'est la même menace qui pèse sur l'agriculture et la sylviculture françaises : à force d'imposer des contraintes nouvelles, de les fragiliser commercialement, nous prenons le risque de voir exploser nos importations ; comme nous avons besoin d'agriculture pour nous nourrir, nous avons besoin de bois pour construire L'abondement de ce fonds stratégique est donc essentiel pour reboiser les forêts en voie de dépérissement, mais aussi pour accompagner les entreprises de transformation dans les investissements qu'elles devront engager afin d'adapter leurs outils aux nouvelles essences, aux nouveaux produits. Cette année encore, le fonds stratégique de la forêt et du bois est amputé des 4 millions d'euros de la taxe affectée plafonnée de défrichement.

Nous comptons sur votre soutien, car la filière mise notamment sur les prochains jeux Olympiques, qui seront l'occasion de promouvoir les usages de matériaux biosourcés dans la construction. Il est également indispensable que le Gouvernement encourage les initiatives privées dans nos forêts. J'ai proposé la création de « certificats de captation carbone », sur le modèle des certificats d'économie d'énergie. Ces certificats pourraient efficacement concourir à la réalisation de l'objectif de neutralité carbone en 2050. présent, le Gouvernement préfère se contenter des démarches volontaires de quelques grandes entreprises ou associations, certes louables, mais tenant plus d'opérations de communication que d'un véritable plan de sauvegarde et de relance de la forêt

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la fin de l'année est marquée, comme en 2018, par un mouvement de contestation de la part de nos agriculteurs. Si la mobilisation semble moins massive cette année, il n'empêche que le malaise paysan demeure toujours aussi profond en France. Les questions fondamentales des revenus agricoles, de l'assurance chômage et des retraites restent pour l'heure sans réponse. Or la plupart de nos agriculteurs vivent dans une grande précarité, qui crée de plus en plus de situations personnelles et professionnelles dramatiques. À cela s'ajoute, chez les professionnels agricoles, le sentiment de ne pas être assez soutenus face aux pratiques de concurrence déloyale déloyale d'autres pays. Nos agriculteurs sont pris en tenaille entre une exigence de qualité exemplaire et une guerre des prix intenable. Dans ce contexte,

avec 3 011,2 millions d'euros inscrits en autorisations d'engagement et 2 957,8 millions d'euros en crédits de paiement. Cette stabilité ne doit pas faire oublier la baisse de 350 millions d'euros des crédits du projet de budget pour 2020 par rapport au budget pour 2018, soit une baisse de 10 %. vient confirmer la tendance à une baisse sensible des crédits agricoles dessinée par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Or c'est précisément aujourd'hui que nos agriculteurs ont besoin de preuves de soutien Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a fixé trois priorités pour le budget de 2020. Première priorité : le soutien aux revenus des agriculteurs, avec la garantie de contreparties nationales à la baisse des aides européennes au titre de la politique agricole commune. Deuxième priorité : la sécurité sanitaire de notre territoire et de nos aliments. Cette exigence répond aux recommandations émises par mes collègues de la commission des affaires économiques dans leur rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2019. C'est d'autant plus important que le Brexit aura des conséquences sur les capacités de la France à contrôler la qualité sanitaire des denrées alimentaires importées. Aussi le budget pour 2020 consacre-t-il la hausse des crédits destinés à lutter contre les maladies animales, ainsi que la création de 320 équivalents temps plein supplémentaires pour renforcer les contrôles sanitaires aux frontières avec le Royaume-Uni. C'est un point positif. Troisième priorité : la formation des jeunes et l'innovation, axe majeur, évidemment, pour l'avenir de notre modèle agricole et pour sa place dans notre économie.

Préparer l'avenir, c'est anticiper la transformation de notre environnement. Les épisodes climatiques de plus en plus extrêmes se multiplient, qu'il s'agisse de sécheresse ou d'inondations. Ces épisodes ont des incidences majeures sur les métiers agricoles et la production. Ce budget ne semble pas faire suffisamment droit à cette réalité ; il est grand temps de prendre la mesure de ces changements et de donner aux agriculteurs les moyens d'y faire face sur le long terme.

Monsieur le ministre, mercredi dernier, les agriculteurs sont venus à Paris crier leur mal-être, souvent leur grande détresse. Que faites-vous pour répondre à leur angoisse ? Vous affirmez régulièrement dans cet hémicycle que vous soutenez nos agriculteurs. J'ai le regret de vous dire, monsieur le ministre, que le projet de budget que vous nous présentez aujourd'hui ne donne pas le signal tant attendu par la profession. Hélas, ce n'est que la suite logique de ce qui s'est passé, par exemple, avec la loi Égalim : beaucoup d'espoir et, malheureusement, à ce jour, pour grand nombre de nos agriculteurs, pas d'amélioration de revenu Vous parlez beaucoup de transition écologique. Là encore, la déception est grande : il n'y a rien dans le projet de loi de finances pour 2020 pour accompagner nos agriculteurs dans une mutation profonde des modes de production de leurs exploitations. Ce texte souffre d'un manque de vision.

En effet, la recrudescence de la tuberculose bovine peut inquiéter. L'essentiel des cas, pour le moment, se concentre en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de foyers a augmenté de 30 % en 2018. Il y a urgence à traiter

les éleveurs de porcs soufflent. Cette embellie ne sera peut-être pas durable. Eu égard aux nombreux défis qu'ils doivent relever, le renforcement de leur compétitivité passe par des investissements. Comment l'État peut-il leur donner un signal fort pour qu'ils profitent de ce haut de cycle pour investir ? Je soutiens, à cet égard, la solution adoptée par le Sénat lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, qui permettra aux éleveurs de suramortir leurs investissements et ainsi de renforcer leur résilience, de réduire l'usage d'intrants ou de veiller à la santé et au bien-être des animaux.

De telles contraintes peuvent les dissuader de s'engager dans le processus de l'installation. Pourtant, cette démarche permet d'avoir des projets sûrs, cohérents et durables. trouver une solution pour remédier à cette situation ? Les chambres d'agriculture ont fait des propositions en la matière. Peut-on envisager qu'elles soient examinées ? Notre agriculture relève aujourd'hui d'un choix de société votre politique ne me paraît pas à même de relever ce défi. Notre indépendance alimentaire est en jeu. C'est pourquoi, comme nombre de mes collègues, je ne voterai pas les crédits pour 2020 de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

pour y parvenir. Veiller à l'unité de nos territoires, c'est d'abord refuser la stigmatisation de nos paysans, comme vous avez été nombreux à l'exprimer à cette tribune. Au risque de me répéter, je veux dire de nouveau ici, au nom du Gouvernement et en mon nom personnel, que les agriculteurs ne sont ni des empoisonneurs ni des pollueurs.

odeurs, nos agriculteurs ne peuvent pas le comprendre. Mais que faites-vous ? Monsieur Bizet, vous qui êtes président de la commission des affaires européennes et qui avez une haute

Actuellement, nos agriculteurs et nos entreprises sont en passe de relever le défi gigantesque de nourrir la population, qui augmente, tout en promouvant la transition agroécologique. Telle est la transition qu'est en train de réussir l'agriculture en France : contribuer à l'autonomie alimentaire, continuer à nourrir la population, tout en progressant vers la transition agroécologique. L'alimentation issue de notre agriculture est de grande qualité.

Trouvez un autre budget qui augmente en 2020 de plus de 9 % ! Les filières ultramarines, oubliées dans la discussion, ont été spécifiquement prises en compte, avec un soutien de 179 millions d'euros. Je pense, notamment, au maintien de l'aide exceptionnelle au sucre,

Nous renforçons les moyens dédiés aux mesures agroenvironnementales et climatiques, ainsi qu'à la conversion à l'agriculture biologique, en vue d'atteindre l'objectif de 15

Veiller à l'unité de nos territoires, c'est aussi rémunérer décemment ceux qui nous nourrissent. Vous l'avez souligné à plusieurs reprises, personne d'autre n'accepterait de travailler autant sans pouvoir vivre de son travail.

contrats d'objectifs et de moyens qui doivent être mis en place. Enfin, veiller à l'unité de nos territoires, c'est faire preuve de solidarité quand les intempéries et la sécheresse frappent.

pour aléas, si j'avais pu ne mettre que 100 millions d'euros, je l'aurais fait. Je ne confonds pas la comptabilité et les orientations politiques. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est inscrit en comptabilité publique, c'est ce qui est effectivement versé aux agriculteurs

Brexit. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai voulu concentrer mon propos sur ce qui m'apparaît être au coeur du projet de réconciliation des territoires. Je pense que ce budget peut permettre d'aider l'agriculture à s'en sortir. Certes, il n'y suffira pas : il faudra aussi que la société change,

de consommateurs. Mesdames, messieurs les sénateurs, je regrette que vous ne soyez pas plus nombreux à vouloir voter ce projet de budget. J'espère néanmoins que nous nous retrouverons, quelle que soit l'issue du vote, pour faire en sorte que l'agriculture de demain soit la plus résiliente possible et, surtout,

Nous devons être « capables de coexister avec notre puissance », comme le dit Hubert Reeves. Nous sommes face à une situation inédite dans l'histoire de l'humanité, l'enjeu ultime étant notre existence même en tant qu'espèce, menacée comme les autres. L'important est non pas d'être optimiste ou pessimiste, mais déterminé, et d'enclencher des politiques volontaristes en révisant nos actions à l'aune des changements nécessaires.

Les maires sont de plus en plus nombreux à prendre des arrêtés interdisant l'utilisation des pesticides à moins de 150 mètres des habitations et 96 % de nos citoyens soutiennent cette démarche ; il s'agit de répondre à ces attentes. Cela relève du principe de précaution.

Nous nous devons d'apporter des réponses concrètes. Faisons confiance aux agriculteurs pour inventer l'agriculture de demain

organiser une concertation entre les agriculteurs et les riverains, demander aux agriculteurs d'ouvrir leur ferme et d'expliquer leur métier, et aux riverains de participer à la vie agricole de leur village. Ce serait bien plus bénéfique

afin de favoriser la transition agroécologique et alimentaire et l'adaptation de la restauration collective à une alimentation de qualité. La loi Égalim a permis une avancée en fixant des objectifs d'au moins 50

de construire des circuits d'approvisionnement locaux en lien avec les acteurs du territoire, de sensibiliser les personnels afin qu'ils changent leurs habitudes, de réaliser des diagnostics, notamment sur le gaspillage alimentaire,

De nombreux groupes politiques et syndicats agricoles avaient demandé que cet organisme public fixe les indicateurs de coûts de production cette demande avait été relayée par le biais de plusieurs amendements. Le Gouvernement et le rapporteur s'y étaient opposés et avaient fait le choix d'attribuer ce rôle aux interprofessions, au sein desquelles existe pourtant un rapport de force déséquilibré. dans la pratique, cette loi n'a absolument pas eu l'effet escompté et n'a pas permis de garantir un meilleur revenu aux agriculteurs. D'ailleurs, les derniers chiffres publiés par l'association UFC-Que Choisir montrent que les relations commerciales ne se sont pas rééquilibrées et que le relèvement du seuil de revente à perte n'a pas conduit à un ruissellement vers les paysans, qui ne vivent toujours pas mieux. Afin que l'OFPM puisse mener à bien ses missions, particulièrement en matière d'aide à la détermination des coûts de production, il est souhaitable de lui allouer des moyens supplémentaires, notamment pour augmenter ses effectifs. Afin de rendre cet amendement recevable,

en transférant 10 millions d'euros du programme 149. Cela conduirait à réduire les moyens dédiés à la modernisation des exploitations agricoles, ce qui ne paraît pas acceptable à la commission des finances.

l'avis du Gouvernement ?

Monsieur le ministre,

de donner au CNPF les moyens dont il a besoin pour mener son action.

Nous prenons acte de cette situation et souhaitons vivement que ses crédits soient rétablis.

monsieur le ministre,

Madame la sénatrice, je salue votre constance ! Je connais votre engagement sur ce sujet. Encourager les étudiants vétérinaires à s'installer en zones rurales et ainsi lutter contre la désertification vétérinaire

Qui plus est, siègent en son conseil d'administration, outre l'État, des représentants des collectivités territoriales et des chambres d'agriculture ultramarines, ce qui en fait une instance de dialogue et de recherche du consensus sur la politique agricole mise en oeuvre. l'Odéadom a fortement contribué, ces dernières années, à orienter l'agriculture des outre-mer vers la diversification. Cela ne pourrait plus être le cas à l'avenir si seules les grandes exploitations et les grandes filières pouvaient constituer des dossiers structurés, alors que l'Odéadom remplit aujourd'hui un rôle d'orientation et de conseil utile et concret. Enfin, le Gouvernement, qui milite pour le développement de circuits courts et la production locale, en le supprimant d'un opérateur efficace, expert signalé des filières agricoles et aquacoles pour l'outre-mer. Cet amendement a pour objet

monsieur le ministre.

II-687 rectifié. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite.